chers collègues, M. Jean Noël Guérini a fait connaître au président du Sénat qu’il démissionnait de son mandat de sénateur des Bouches du Rhône à compter du mercredi 20 mars 2024, à minuit. En application de l’article L.O. 320 du code électoral, il a été remplacé par Mme Mireille Jouve, dont le mandat a commencé ce jour, à zéro heure. Écologiste – Kanaky, la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et

l’examen, par le Sénat, du projet de loi autorisant la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada – le (Ceta) – ainsi que de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Canada nous offre l’occasion de faire le bilan de deux accords provisoirement en vigueur depuis bientôt sept ans. Je veux l’affirmer d’emblée, très clairement, avec force et sans ambiguïté ces deux accords sont bons pour notre économie, pour nos entreprises, pour notre agriculture et pour notre relation stratégique avec le Canada. Les débats enflammés sur le Ceta et le flot de contrevérités qui ont circulé ces derniers jours nous ont presque fait oublier que nous avions à discuter aujourd’hui de deux accords.

L’Union européenne et le Canada, ce sont deux piliers dans un monde qui perd ses repères. L’Union européenne et le Canada, ce sont deux garants de l’État de droit ; deux défenseurs de la démocratie, des droits humains et sociaux ; deux accélérateurs de notre indispensable transition énergétique. L’Union européenne et le Canada, ce sont deux entités qui partagent des valeurs et des intérêts, et qui doivent, au nom de ces valeurs, maintenir et consolider les liens qui les unissent. En d’autres termes, ils sont, l’un pour l’autre, un partenaire incontournable. J’ose le dire : pour l’Union européenne, comme pour la France, le Canada est plus qu’un allié. C’est un ami, un partenaire historique. C’est un pays francophone, ce qui est évidemment important pour nous, Français. C’est un partenaire qui, sur le plan des échanges commerciaux, nous offre des perspectives de stabilité de long terme dont nous avons absolument besoin, alors que les impérialismes montent de toutes parts et que les guerres et les tensions géopolitiques perturbent le commerce mondial. Je veux d’abord évoquer l’accord de partenariat stratégique, qui constitue un premier fondement de notre rapprochement avec le Canada. Ces dernières années, outre le travail étroit qu’ils ont réalisé pour soutenir l’Ukraine,

l’Union européenne et le Canada tiennent ensemble un sommet annuel qui permet la mise en œuvre de ces ambitions communes. Cet accord est fondamental, en ce qu’il offre le cadre d’un partenariat de très haut niveau.

Les chiffres parlent d’eux mêmes. Les exportations françaises ont bondi de 33 % en six ans, tous secteurs confondus. C’est d’abord vrai dans le secteur industriel l’exportation de produits chimiques et cosmétiques a augmenté de moitié en l’espace de six ans ; celle des produits sidérurgiques a doublé ; celle des textiles et des chaussures a été multipliée par 2,5. Quant à l’exportation de nos services,

Trop de fausses informations ont circulé sur vos boîtes mail et vos boucles WhatsApp ou Telegram, mesdames, messieurs les sénateurs. Il est temps de rétablir la vérité ! Depuis le Canada, nous n’importons quasiment aucune viande de porc

que, au Canada, ces filières sont loin de pouvoir se structurer pour répondre aux exigeantes règles sanitaires européennes. Nos réglementations européennes et françaises sont strictes. Elles jouent un véritable rôle de garde fous, nous prémunissant contre l’importation de viande traitée aux hormones ou aux antibiotiques utilisés comme facteurs de croissance. Ce sont les fameuses mesures miroirs, monsieur le rapporteur pour

effectue un suivi sanitaire, à la fois au Canada et à l’entrée des produits sur le marché européen, ce qui ne nous empêchera évidemment pas de continuer à travailler avec le Canada et les services sanitaires et douaniers français et européens pour renforcer la qualité des contrôles. Il m’a semblé entendre une autre inexactitude, selon laquelle l’accord serait davantage bénéfique au Canada. Comment serait ce possible, alors que l’accord a massivement profité à nos PME, dont l’internationalisation est une nécessité ? Comment serait ce possible alors que, en plus de l’accélération de nos exportations, l’accord a ouvert à nos entreprises l’accès aux marchés publics canadiens, par exemple dans les secteurs des transports et des énergies renouvelables ? Certes, nous importons depuis le Canada autant que nous exportons.

Quant au pétrole canadien que nous importons, il se substitue au pétrole russe… Bref, dans la politique de diversification des approvisionnements et de sécurisation des accès à ces matières essentielles pour notre souveraineté, nous avons besoin du Canada.

Nous partageons avec le Canada une langue, des valeurs fondamentales, une même conception de la démocratie et de la gouvernance mondiale. Nous partageons avec lui des combats pour les droits humains et sociaux et pour l’environnement.

Mais ai je vraiment besoin de rappeler tout cela devant le Sénat, qui, avec l’Assemblée nationale, la Chambre des communes et le Sénat canadiens, participe, depuis 1965, à l’Association interparlementaire France Canada

commerce. Pour être prospères, nous avons besoin de commerce et nous avons besoin d’exporter. On ne peut pas à la fois se plaindre d’une balance commerciale en déficit et tuer les initiatives qui nous aident à redresser la barre.

Ses règles protègent nos filières et leur permettent d’exporter, d’investir. Surtout, elles ne dérogent à aucun de nos principes environnementaux ou sociaux. Si ! Ce n’est pas le cas de l’accord en cours de négociation avec les pays du Mercosur, raison pour laquelle le Gouvernement s’y oppose et continuera de s’y opposer.

L’histoire a déjà montré que la fermeture commerciale n’est pas une solution pour des économies qui ont besoin, en priorité, d’améliorer leur compétitivité. » Ces propos – vous pourrez le vérifier, monsieur le rapporteur pour avis – ont été tenus par Laurent Wauquiez, en 2011. J’irai plus loin que lui : l’histoire a déjà montré que la fermeture commerciale, le rétrécissement de la mondialisation que représente le protectionnisme font partie des voyants qui s’allument lorsque le monde s’apprête à sombrer. aux élus de droite : ne tombez pas dans le piège d’une alliance incongrue et contre nature avec les communistes, qui vous conduirait à renier vos principes au prétexte de répondre à la colère que peuvent susciter certains autres traités. Mettez la campagne des élections européennes entre parenthèses le temps d’un vote. N’entraînez pas notre pays sur la voie du repli ! La droite sénatoriale, héritière d’une famille politique à laquelle j’ai appartenu t elle qu’elle fut, un jour, le point de rassemblement de ceux qui croyaient en l’Europe, qui défendaient le commerce, qui croyaient en un libéralisme respectueux de notre modèle social ? Non !… La droite sénatoriale s’élèvera t elle contre un texte qui, avant François Hollande, fut négocié par le président Nicolas Sarkozy ? Non !… La droite sénatoriale votera t elle à rebours de l’injonction de celui qui a été l’une de ses plus grandes figures pendant tant d’années, Jean Pierre Raffarin,

Mesdames, messieurs les sénateurs du groupe Les Républicains, ne suivez pas les partisans du repli sur soi et du recroquevillement ! De qui parlez vous ? Aux élus socialistes et écologistes, je veux

N’ajoutons pas une crise aux crises ! J’en appelle à la sagesse qui a toujours caractérisé la chambre haute. Jugeons le réel, et disons « oui » à cet accord

dont fait preuve votre gouvernement non seulement envers le Sénat, mais aussi envers les sénateurs qui ne pensent pas comme vous. Votre déni est consternant – je dirais même « pathétique

Pour autant, nous ne saurions nous réjouir de cette situation, car il nous est demandé – ni plus ni moins – de nous prononcer sur un texte dont près de 90 % du contenu est mis en œuvre depuis près de sept ans.

était juridiquement possible. Mais, alors que chacun connaît la sensibilité des questions agricoles à l’échelle nationale, appliquer provisoirement un tel accord ne revient il pas à mettre les parlementaires nationaux au pied du mur, en considérant qu’ils n’oseront pas le dénoncer parce qu’il produit déjà des effets ? On peut aussi s’interroger sur le caractère démocratique du maintien en vigueur d’un accord qu’un Parlement d’un pays souverain – celui de Chypre – a rejeté.

quitte à passer outre la volonté du Parlement. À quelque chose malheur est bon : cette situation nous permet de juger concrètement des effets du Ceta. Quel bilan pouvons D’abord, l’impact sur le commerce bilatéral semble positif, à l’échelon tant européen que français. Les échanges entre la France et le Canada ont ainsi progressé de 33 % entre 2017 et 2023, passant de 6 à 8 milliards d’euros.

nous avons consommé nos quotas. Derrière ces chiffres répétés à l’envi par les défenseurs du Ceta, à quelle réalité concrète faisons nous face ?

Enfin, et c’est peut être le plus important, une étude économique réalisée par le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii) montre que les effets du Ceta sur la croissance française et européenne

une fois, les défenseurs de l’accord mettront en avant le fait que le Canada sous utilise le contingent de viande bovine dont il dispose.

Par ailleurs, cette situation est loin d’être immuable, pour plusieurs raisons. En premier lieu, une forte dépendance des exportations canadiennes de viande vis à vis des marchés américain et asiatique pourrait conduire les producteurs canadiens à s’intéresser d’un peu plus près au marché européen. L’argument selon lequel un tel scénario ne s’est pas produit en presque sept ans de mise en œuvre n’est pas recevable : chacun peut comprendre la frilosité des producteurs canadiens à consentir des investissements importants en Europe, alors que le Ceta n’est pas définitivement adopté. En second lieu, et c’est peut être là l’essentiel, si les autorités européennes devaient céder aux demandes canadiennes

Compte tenu des différences fondamentales entre les modèles d’élevage européen et canadien, nos éleveurs ne pourraient pas faire face à la montée de la concurrence canadienne Plus généralement, nous ne pouvons que regretter que la Commission européenne négocie des accords dépourvus de clauses miroirs, c’est à dire sans réelle réciprocité des normes.

Certes, l’application de l’accord ne conduit pas à revoir nos normes, mais les réglementations applicables aux importations depuis des pays tiers diffèrent de celles qui s’imposent à nos agriculteurs.

pour le respect d’un principe simple : si c’est interdit pour nos agriculteurs, ça ne doit pas rentrer chez nous ». Dont acte ! Commençons par revoir les accords de libre échange qui imposent précisément une telle forme de concurrence déloyale.

le respect de la réglementation européenne par les produits importés suppose l’existence de dispositifs de contrôle efficaces. Or, du côté européen comme du côté canadien, ceux ci souffrent de lacunes côté européen, le Ceta prévoit un abaissement du taux de contrôle physique dans les postes d’inspection aux frontières ; côté canadien, à l’occasion d’un audit mené en 2019, la Commission européenne a relevé des défaillances dans le système de contrôle et de traçabilité, et un second audit, conduit en 2022, a mis en évidence la persistance des lacunes constatées trois ans plus tôt.

en matière de bien être animal et de renforcement de notre souveraineté alimentaire. C’est pourquoi la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté un amendement visant à supprimer l’article 1 du présent projet de loi, c’est à dire à refuser la ratification de l’accord économique.

Je sais bien que, de l’autre côté de l’Atlantique, ce rejet pourra surprendre ou décevoir. Je veux dire avec force qu’il ne devra pas être interprété comme un rejet du Canada,

Voilà déjà cinq ans que nous aurions dû nous prononcer sur la ratification du Ceta, si le Gouvernement n’avait pas eu peur de le soumettre au Sénat.

S’il est vrai que les premières années ont été fructueuses, depuis quatre ans, les choses se sont inversées et augurent de la suite. Savez vous que la balance commerciale de la France avec le Canada est déficitaire, cette année, de 23 millions d’euros ? le Gouvernement a fait sien le mot de Churchill : il ne croit aux statistiques que lorsqu’il les a lui même falsifiées. Pour prouver cela, tout est bon

Cepii, un service du Premier ministre, la révèle : cet accord fera augmenter nos importations trois fois plus vite que nos exportations. En tout et

an par Canadien. Voilà la seule contrepartie du lourd tribut que nous allons payer en renoncements, en reniements et en naïveté coupable d’une Commission européenne engluée dans ses contradictions ! Je vous le dis tout net nous ne pouvons plus continuer à importer d’ailleurs ce que nous interdisons de produire chez nous. Nous devons dire « stop » – et nous allons le faire ! – à la concurrence déloyale que nous faisons subir aux producteurs européens de tous ordres, agricoles et non agricoles, en imposant des normes toujours plus draconiennes chez nous tout en fermant les yeux sur les produits importés. Comment expliquer, monsieur le ministre, le silence de la Commission européenne après les deux audits qu’a réalisés, au Canada, en 2019 et 2022, sa direction générale de la santé, qui constataient des lacunes sur la traçabilité animale ne permettant pas de garantir du bœuf sans hormones ? de nos frontières, nous interdisant d’exporter. Comment pouvons nous collectivement, nous les Européens, faire preuve d’une telle naïveté coupable en nous comportant comme des tigres avec nos producteurs européens et comme des agneaux avec les Canadiens ? Comment avons nous pu céder à chaque fois aux demandes de dérogation faites par les Canadiens ou bénéficiant au Canada ? En 2013, nous avons accepté, dans le cadre des négociations avec le Canada et les États Unis, l’utilisation de l’acide lactique pour la décontamination des carcasses. En 2018, le Parlement européen a voté une mesure miroir interdisant l’utilisation d’antibiotiques

un simple certificat sur l’honneur signé par un vétérinaire sur place. Que va faire la Commission de la dernière demande de dérogation de décembre 2023 pour l’utilisation de l’acide peracétique afin de décontaminer les carcasses ? Je vous le dis : elle cédera, comme elle l’a toujours fait ! Ainsi, votre seul argument, monsieur le ministre,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

L’Assemblée nationale s’étant prononcée en juillet 2019, le Sénat attendait depuis de longues années de pouvoir traiter le sujet. En 2021, à la suite de l’adoption d’une résolution déposée par notre collègue Fabien Gay, 309 sénateurs appelaient de leurs vœux l’inscription de ce projet de ratification à l’agenda sénatorial. Monsieur le ministre, nous n’en serions pas là aujourd’hui si le Gouvernement avait daigné entendre cet appel à débattre démocratiquement, dans le respect dû à notre chambre. L’avis du Sénat, toujours constructif, sait être utile, voire salutaire à l’exécutif. Sept ans après l’entrée en application provisoire de près de 95 % des termes du Ceta, le temps est venu, à n’en pas douter, d’engager le dialogue,

Mes chers collègues, je veux vous convaincre du bien fondé de cette motion de procédure, dont l’objectif n’est pas le renvoi de ce texte aux calendes grecques, mais bien son examen précis, comme notre assemblée sait si bien le faire.

Le 21 septembre 2017, près de 95 % des mesures du Ceta sont entrées en application provisoire, car elles relevaient des compétences exclusives de l’Union européenne en matière de droits de douane et de politique commerciale. Si les Parlements sont sollicités pour une ratification, c’est parce qu’il s’agit d’un accord dit de nouvelle génération, dont 5 % des termes relèvent des compétences partagées de l’Union européenne avec les États membres, et non de ses compétences exclusives.

Éclairons le débat, sans emprunter les raccourcis vers lesquels veut nous mener la campagne de désinformation massive sur le Ceta ! Sur le plan stratégique, le Canada est un partenaire de premier ordre pour notre pays. Nos liens d’amitié sont anciens, nos cultures et nos visions stratégiques sont proches, nous partageons des valeurs similaires sur les droits humains et sociaux, sur l’État de droit ou encore sur la gouvernance mondiale.

Nous développons une coopération sectorielle renforcée en matière de climat, d’environnement et de diversité culturelle. La coopération universitaire et en matière de recherche innovation est particulièrement dynamique, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’une des priorités affichées de la politique – extérieure comme intérieure – canadienne est la lutte contre le changement climatique, tout comme chez nous. Le Canada n’est pas un loup d’Alberta, un prédateur ; il est un ami, un allié de la France.

des amalgames, mes chers collègues. J’en viens à présent à la forme. En premier lieu, la tenue de ce débat dans le contexte des élections européennes du 9 juin prochain apparaît comme une opération montée de toutes pièces, une mauvaise pièce de théâtre où le rideau de fin tombe avant les trois coups. En outre, le débat sur la ratification du Ceta ajoute de l’huile sur le feu aux vives tensions que connaît le monde agricole. Tout cela vient brouiller notre nécessaire prise de recul, pour ne nourrir nos discussions que de postures politiques.

à nos entreprises, avec une augmentation des exportations de plus d’un tiers entre 2017 et 2023, et notre marge de progression est encore grande. Le secteur des services a connu une hausse de ses exportations de 71 %.

Les débouchés pour nos entreprises sont donc bien réels. Les échanges depuis le Canada vers la France sont eux aussi essentiels pour nos entreprises. Ils nous permettent de nous approvisionner en métaux critiques – uranium, titane, zinc, lithium, potasse, graphite –, minerais nécessaires à nos secteurs industriels clés et à la mise en œuvre de notre politique de transition écologique. Quant aux importations de pétrole canadien, elles contribuent tout simplement à réduire notre dépendance énergétique envers la Russie. Mes chers collègues, Mes chers collègues, faisons un focus sur le secteur agricole, principale préoccupation de nombre d’entre nous. Les bénéfices sont, là aussi, réels : l’excédent des filières agricoles et agroalimentaires a été multiplié par trois

Les rapporteurs nous ont présenté leurs travaux, réalisés dans un temps record et contraint, mais de nombreuses questions subsistent avant de pouvoir dresser un bilan objectif du Ceta : avons nous une idée de ses impacts sur nos PME et autres

Et, face à nos concitoyens, aurons nous le courage de nos positions, lorsque nos filières fromages et vins verront leurs exportations chuter en raison de la mise en place de nouvelles barrières douanières ? Les assumerons nous quand il s’agira de justifier le manque de diversification de nos sources d’approvisionnement en minerais nécessaires à à nos différentes industries, dont nous prônons la souveraineté ? Quel message serait envoyé à notre cousin et allié canadien, avec lequel nous consolidons des relations stratégiques ? Quel signal

Avons nous interrogé nos partenaires européens à ce sujet ? À toutes fins utiles, je rappelle que le Ceta reste un accord dynamique, qui prévoit des dispositions de révision. Usons de notre sérieux pour travailler ensemble à ces améliorations et demandons nous aussi des garanties Pour conclure, tant sur le fond que sur la forme, la position précipitée de notre assemblée sur ce texte nous porterait un discrédit sans précédent. Mes chers collègues, chacun de nos prédécesseurs, chacun d’entre vous a contribué à asseoir le sérieux des travaux du Sénat. Ne sacrifions pas le Ceta sur l’autel des postures politiques. Laissons ce loisir à d’autres, et conservons notre image de sérieux en votant cette motion de procédure, dont l’objectif unique est de permettre un travail au fond. Nous attendions tous ce moment,

Pour qu’il soit serein, il faut, monsieur le ministre, que le Parlement soit respecté. Pour qu’il soit approfondi, mes chers collègues, nous avons fait le choix d’annoncer, dès le début du mois de février

De plus, l’argument selon lequel l’inscription de ce texte dans une niche parlementaire ne permettrait pas un examen en profondeur n’est pas recevable. J’estime, pour ma part, que, avec plus de cinq ans,

Depuis 2019, année au cours de laquelle le projet de loi a été déposé, le monde a beaucoup changé. C’est pourtant du même texte que nous discutons aujourd’hui, dans le cadre d’une niche parlementaire. Que souhaitons nous obtenir par un vote négatif ? Remettre en cause le futur accord du Mercosur ? Ce projet est totalement disjoint du Ceta et de la discussion que nous avons aujourd’hui. Obtenir de meilleures garanties lors d’une éventuelle rediscussion de l’accord ? Lesquelles ? Et avec quels alliés en Europe ? Je vous le redis, mes chers collègues : en votant contre le Ceta, nous remettrions en cause un accord qui est considéré, dans de nombreux secteurs économiques, comme indispensable et bénéfique pour l’Europe. Évidemment ! En votant contre le Ceta, nous affaiblirions la position française dans toute future négociation commerciale. En votant contre le Ceta, nous remettrions en cause nos relations avec un allié historique qui ne nous a jamais fait défaut. Je constate aujourd’hui que les conditions permettant la tenue d’un

dix ans de négociations pour aboutir à un accord, en 2016. Durant ces dix années, les parlementaires ont eu la possibilité de s’intéresser

commis un véritable déni de démocratie. Nous vous appelons donc solennellement, monsieur le ministre, à ne pas prolonger ce mauvais traitement, en permettant que la navette parlementaire se poursuive, et, en cas de rejet du Ceta, à le notifier à la Commission européenne, par respect pour nos institutions et pour nos concitoyens. J’en viens au contenu de l’accord. La Commission européenne, relayée par le Gouvernement, met en avant, dans sa communication, une évolution importante des échanges, en omettant de préciser qu’il s’agit d’une augmentation en valeur non retraitée de l’inflation, ce qui diffère sérieusement de l’évolution en volume, estimée par Eurostat à seulement 0,7 point entre 2017 et 2022, attestant l’effet marginal de l’application provisoire du Ceta. De même, les partisans de l’accord soulignent l’évolution de secteurs d’activité, qui profiteraient de la disparition des barrières tarifaires, comme le textile, les vins et spiritueux ou les fromages, mais ces secteurs restent marginaux dans notre balance commerciale. On essaie aussi d’apaiser les craintes de nos agriculteurs sur les importations de viande bovine, le Canada n’ayant quasiment pas utilisé ses quotas. Devons nous cependant être rassurés quand les animaux sont nourris avec de la farine animale, que le Canada a obtenu des dérogations aux normes européennes sur la décontamination des carcasses et que les audits de la direction générale

davantage sur le volet agricole, sur lequel mon collègue Jean Claude Tissot reviendra. Outre les barrières tarifaires et non tarifaires, cet accord porte sur un large champ d’intervention, incluant notamment la libéralisation des services publics, jusqu’alors protégés. Le Ceta est, par ailleurs, en totale contradiction avec nos engagements environnementaux. Alors que l’article 2 de l’accord de Paris engage les pays signataires à limiter l’extraction et le commerce d’énergies fossiles par des restrictions d’importations, ces derniers représentent 40 % des échanges visés

qui contribuent à des émissions massives de gaz à effet de serre et sont fortement carbonés. Nous sommes loin de l’image idyllique que l’on nous présente… Si l’accord de Paris et la protection de l’environnement sont évoqués dans la déclaration interprétative, rien ne les rend opposables ni juridiquement contraignants.

Six ans plus tard, les résultats l’attestent : les promesses du Gouvernement d’éviter ces effets négatifs se sont évaporées. La commission Schubert avait aussi alerté sur la création d’une coopération réglementaire, dont est « la plus préjudiciable à l’autonomie des parties contractantes dans l’élaboration de leur réglementation ». Rappelons le, l’accord a pour finalité d’éliminer les obstacles au commerce et aux investissements instaurant la prééminence du droit commercial sur tous les autres, devant la protection de l’environnement, devant la protection des consommateurs et devant la protection des travailleurs. dispositions du Ceta sont appliquées, nous sommes appelés à ratifier cet accord de caractère mixte, car il inclut un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. Cela constitue, à nos yeux, un outil supplémentaire pour que les multinationales puissent contester et peser sur les décisions des États souhaiteraient instaurer des normes environnementales et sociales plus protectrices. Ce système, s’il était validé, leur permettrait d’attaquer les États ou l’Union européenne dès qu’elles considéraient qu’une réglementation nuirait à leur activité. Même si les États ne seront pas contraints de modifier leur réglementation, cela représente une menace,, sur l’édiction des normes, et,, sous la forme de dommages et intérêts exorbitants. Enfin, dernière incongruité, la France vient de sortir du traité sur la Charte de l’énergie, qui protège les investissements dans les énergies fossiles. Or le Ceta octroie à ces investissements une protection juridique de même nature que le traité, en

que ce soit les 100 000 tonnes de blé, les 8 000 tonnes de maïs doux, les 75 000 tonnes de viande de porc ou encore les 48 000 tonnes de viande de bœuf, sont, en réalité, issus d’une tout autre agriculture. Loin des standards européens et français, l’agriculture du centre du Canada, de l’Alberta par exemple, est jumelle de celles du Brésil, de l’Argentine ou des États Unis, aux antipodes de notre modèle d’exploitation familiale. Plus de

Vous avez parlé des lentilles vertes du Puy, monsieur le ministre. Le glyphosate, par exemple, est utilisé de façon récurrente pour accélérer la maturité des lentilles au Canada, jusqu’à quatre jours avant la récolte. L’Europe interdit cette pratique. Nous

sans identification individuelle de l’animal, sans garantie sur la qualité indemne du cheptel, comme cela existe en France. La logique qui prévaut est de s’affranchir des règles sanitaires contraignantes tout au long de la vie de l’animal et d’effacer le risque sanitaire en fin de cycle, à l’abattage, par la décontamination des carcasses à l’acide.

le disent : « Nous avons le droit de réglementer dans notre pays souverain de la manière que nous jugeons appropriée et adaptée à notre environnement local. »

réaffirmerons ainsi nos liens si importants avec le Canada, dans le respect de nos producteurs français et européens. La parole est à M. Stéphane Ravier.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce n’est pas pour rien que la gauche socialiste, emmenée par un certain François Hollande, a soutenu le Ceta. Le libre échange avec l’extérieur de nos frontières est, en effet, l’ennemi de la libre entreprise à l’intérieur. La Commission von der Leyen, fidèle à celle de Juncker, cherche à libéraliser les échanges à l’extérieur de l’Union, tout en submergeant de contraintes les entrepreneurs des mêmes secteurs européens et français. Pour nos paysans, cela revient à moins de compétitivité pour plus de compétition. La mondialisation économique heureuse n’existe pas : il y a des gagnants et des perdants. Nous sommes des perdants consentants ! Non seulement vous avez fait de nous des cocus, mais vous exigez, en plus, que nous soyons contents, J’en veux pour preuve que le Ceta supprime 98 % des droits de douane sur les importations canadiennes, quand, dans le même temps, le Pacte vert européen ajoute soixante quinze lois pour administrer l’agriculture à la parcelle près. Dans ce contexte, le méga éleveur canadien est un concurrent déloyal pour le paysan français. La transition écologique de Bruxelles est une transition du déficit. Depuis la mise en œuvre partielle du traité en 2017, le déficit commercial de la France avec le Canada s’établit non pas à 23

Un échange sans réciprocité n’est pas un libre échange. Pendant que nos agriculteurs sont surveillés par drone et visités par les agents armés et impitoyables de l’Office français de la biodiversité, une simple attestation sur l’honneur exempte l’exportateur canadien de tout contrôle et de droits de douane. Pourtant, au Canada, le bœuf est engraissé dans des fermes industrielles aux milliers de vaches, sans traçabilité. Il est nourri aux farines animales, les mêmes qui causèrent la vache folle. Des antibiotiques peuvent être utilisés comme activateurs de croissance. L’accord prévoit ainsi que 65 000 tonnes de viande de piètre qualité pourront inonder notre marché – autant de viande de qualité que nos éleveurs bovins ne vendront plus ! Le Ceta, c’est

Les perdants seront notamment les filières du maïs doux, des légumineuses et de la moutarde. Par les nombreux accords de libre échange, notamment les accords signés avec le Mercosur et la Nouvelle Zélande, vous court circuitez les circuits courts, Le refus de la ratification du Sénat sera, pour nous, le refus de ce libre échange kolkhozien par lequel l’agriculteur n’est plus qu’un ouvrier de la Commission européenne, devenue maîtresse des cheptels et des moissons. Nous voulons des barrières douanières qui protègent la libre entreprise sur notre sol et garantissent que nous mangions du poulet du Maine plutôt que d’Ukraine, des pommes d’Occitanie plutôt que du Chili, du bœuf de Lozère plutôt que de Vancouver : la Corrèze avant le Zambèze, mes chers collègues, encore et toujours ! Nous voulons une Europe puissance plutôt qu’une Europe nuisance qui sacrifie l’agriculture sur l’autel de la concurrence,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, aujourd’hui, les paysans vont mal, et ce n’est pas nouveau. Aujourd’hui, les paysans vont mal dans toute l’Union européenne, et ils manifestent partout. Surtransposition, non respect des normes sanitaires d’élevage par certains pays européens, coût de la main d’œuvre déséquilibré, importations de blé dur russe, entré en Europe par la Turquie… Hélas ! la liste est longue, et même très longue. Le ras le bol du monde agricole et sa perte de compétitivité, c’est tout ça ! La colère est légitime face à cette triste réalité. Balayons déjà devant notre porte entre États membres ! Nous ne sommes pas condamnés à l’impuissance.

Toute filière d’importation doit être construite et contrôlée par l’Europe avant l’arrivée d’un kilo de viande sur le territoire, d’où qu’elle vienne. Disons le clairement le bœuf aux hormones sur le territoire européen n’est pas possible aujourd’hui et ne le sera jamais. Mais certains, chez nous, préfèrent jouer sur une peur, celle d’un hypothétique futur grand remplacement du bœuf français par du bœuf canadien. De manière pernicieuse, une coalition s’est formée pour associer le Ceta au Mercosur. Or le Ceta n’est pas le Mercosur. Nous

C’est l’export de fromages français, de spiritueux, de vins à haute valeur ajoutée pour nos producteurs et pour les consommateurs canadiens. C’est Alstom, qui a rénové le métro de Montréal et qui équipera demain le Grand Toronto de trains de banlieue, pour 118 millions de dollars. C’est l’importation de minerais stratégiques, qui réduit notre dépendance aux régimes autoritaires et dont notre souveraineté dépend. Qui, dans cet hémicycle, préfère importer des minerais ou du pétrole de la dictature de Poutine plutôt que de nos amis canadiens ? souhaitent fermer les frontières et se replier sur eux mêmes, assumons d’être ouverts sur le monde et de commercer avec des partenaires de longue date.

c’est le paysan qui vous parle, l’éleveur de vaches limousines ! Après le vote, il y aura ceux qui auront fait le choix de l’émotionnel et de l’opportunisme, en utilisant le Ceta pour souffler sur les braises des souffrances des éleveurs, des éleveurs, et il y aura ceux qui auront fait le choix du pragmatisme économique et de la cohérence avec leurs convictions politiques.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je remercie le président Marseille et mon groupe Union Centriste de me faire l’honneur de défendre aujourd’hui, devant vous, le choix de la majorité d’entre nous de ratifier le Ceta, cet accord de libre échange entre le Canada et l’Union européenne. compétence exclusive de l’Union européenne, cet accord est provisoirement entré en vigueur le 21 septembre 2017. Près de sept ans plus tard, comme le ministre l’a brillamment rappelé, son bilan se révèle très positif pour l’Union européenne et pour la France

Le Canada est devenu un partenaire majeur pour notre souveraineté énergétique. Il nous facilite l’accès à des minéraux stratégiques présents sur son sol, sans droits de douane. La chambre de commerce France Canada rappelle que cet accord a permis de créer un espace économique sûr entre l’Europe et le Canada, avec des règles du jeu transparentes, stables et prévisibles.

l’Autriche, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays Bas, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, la Suède et la Roumanie. À écouter nos rapporteurs, il faudrait rejeter le Ceta, en refusant de le ratifier aujourd’hui. Le Sénat n’a pas la capacité de faire tomber le Gouvernement. A t il la capacité d’annuler un accord européen déjà ratifié par l’Assemblée nationale et par deux tiers des pays européens ? La démocratie, ce n’est pas une minorité qui impose sa volonté ! Très bien ! Bravo ! Ne pas ratifier le Ceta aujourd’hui aura surtout pour effet de discréditer notre pays auprès du Canada et de l’affaiblir sur la scène européenne. est la volonté du groupe CRCE K, car les communistes sont contre le libre échange, qui serait, d’après eux, à l’origine d’une « mondialisation malheureuse » pour les peuples. Casser la mécanique européenne fait partie de leur logiciel, comme de celui de l’extrême droite. Ce n’est pas nouveau. Le revirement

Le président du groupe d’amitié France Canada est dans leurs rangs. Quelle honte ! Jacques Delors, réveille toi, ils sont devenus fous ! À l’image de M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, nos rapporteurs s’essaient au trumpisme.,

L’accord devient ici un bouc émissaire, bon pour l’abattoir. Pour vivre en Angleterre, je connais ces tirades démagogiques et anti européennes, qui s’appuient sur la désinformation. Ce sont celles des Brexiteurs Nos collègues républicains, qui vont s’allier aux communistes, pensent qu’ils pourront capitaliser sur les tensions du monde agricole lors du prochain scrutin européen. Ce faisant, ils trahissent tous ceux qui bénéficient du Ceta. Ils trahissent également les présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy,…

Voilà cinq ans que nous demandons que cesse ce hold up démocratique. Questions écrites, résolutions, interpellations… C’est à croire que votre gouvernement a peur du Parlement, ministre ! Je n’oserais y penser… Négocié sous Nicolas Sarkozy, poursuivi sous François Hollande, adulé par Emmanuel Macron : il en aura fallu du temps pour percevoir les effets délétères de ce traité Pour nous, le cap a toujours été clair : cela fait dix ans que les écologistes, dont mon collègue Yannick Jadot, se battent contre les aberrations de ce traité. Pourtant, c’est la première fois que notre chambre en est réellement saisie. Quelle hérésie démocratique ! Depuis plus de six ans, ce traité de libre échange impliquant près de 500 millions de personnes s’applique à 90 %, alors même que dix pays de l’Union européenne, dont la France, ne l’ont pas ratifié. Pire, nous ne savons même pas si un rejet de cet accord entraînera réellement une dénonciation de celui ci par le Gouvernement. Un tel mépris du Parlement sur un sujet aussi important est inacceptable. Mais, puisque cet accord s’applique, tirons en un premier bilan. C’est ce qu’a fait l’Institut Veblen en janvier dernier. La conclusion est sans appel : le Ceta est une catastrophe pour le climat, la santé humaine et la souveraineté des États. Comme tant d’autres accords de libre échange, il soumet notre économie à une concurrence déloyale, particulièrement en matière agricole, et il inféode la France à la loi des multinationales. le bilan économique. Alors que la Commission européenne nous promettait de vastes débouchés à l’exportation et 700 000 emplois soutenus par les exportations vers le Canada, les données disponibles montrent une tout autre réalité. Selon Eurostat et la direction générale au commerce de la Commission européenne, la part des emplois européens liés aux exportations est globalement stable, à l’échelon tant européen que national. Il en va de même pour la part touchant les PME, alors que les négociateurs leur avaient fait miroiter de vastes marchés. Seuls quelques secteurs tirent leur épingle du jeu à l’export, comme l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique et le nucléaire. qui est des importations, nous achetons deux fois plus d’engrais au Canada qu’avant l’entrée en vigueur de l’accord, et les achats de minerais ont également fortement augmenté. Pourtant, certains Surtout, les importations de pétrole issu de schistes bitumineux, c’est à dire issu de sable visqueux, ont augmenté de 50 %. Rappelons que ces hydrocarbures sont trois à quatre fois plus polluants que le pétrole conventionnel, et que leur extraction consomme une quantité astronomique d’eau et de produits chimiques L’exploitation de cette ressource est une véritable barbarie environnementale : des forêts entières sont rasées ; des lacs, des cours d’eau et des rivières sont pollués à jamais. En 2020, devant la Convention citoyenne pour le climat, le Président de la République lui même s’est dit prêt à abandonner le Ceta si celui ci ne respectait pas l’accord de Paris. Il faut maintenant passer de la parole aux actes Sur le volet agricole, cet accord est l’exemple parfait de la concurrence déloyale dénoncée par les agriculteurs. Comme l’indique le rapport Schubert remis en 2017 au Gouvernement, dont les conclusions restent valides, le Canada continue d’autoriser nombre de pratiques interdites ou plus limitées en Europe. Le bétail est ainsi couramment alimenté avec des farines animales, cause possible de la maladie de la vache folle, ou bien avec du maïs et du soja génétiquement modifiés. Les quantités de résidus de pesticides sont également bien supérieures aux seuils autorisés sur notre continent. C’est le cas pour la filière légumineuse, particulièrement touchée par la fin des droits de douane. L’usage des antibiotiques, facteur de croissance, est généralisé, au mépris du bien être animal et de la lutte contre l’antibiorésistance.

miroirs. Parlons en ! Pour l’instant, c’est surtout le Canada qui fait pression pour que nous baissions nos standards. Il a porté plainte devant l’OMC, en 2019, contre les nouvelles règles européennes sur les pesticides et, en 2023, contre l’interdiction des produits contenant deux néonicotinoïdes interdits en Europe. Puis, toujours en 2023, il a demandé un report de l’interdiction d’importation du bétail gavé aux hormones de croissance. Enfin, une ratification du Ceta entraînerait l’application de son dernier volet, peut être le plus dangereux, celui de la protection des investissements, qui permet à des multinationales s’estimant lésées par une loi d’attaquer un État devant un tribunal d’arbitrage privé. Ces recours viennent notamment de groupes engagés dans les énergies fossiles, contre des décisions de fermeture de centrales à charbon ou de fermeture de forages d’hydrocarbures. la menace des amendes peut conduire les États à renoncer à changer leurs lois jusqu’à vingt ans après la sortie de l’accord, en vertu d’une clause de survie. Alors, loin des caricatures, monsieur le ministre,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, enfin !

après sept longues années d’attente, le Sénat va enfin pouvoir se prononcer sur le projet de ratification de l’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne. Mes chers collègues, cela est déjà une première victoire démocratique pour notre assemblée.

car nous refusons ce déni démocratique. Ce traité, imaginé dans les années 1990, négocié en toute opacité dans le troisième sous sol de la Commission européenne pendant une décennie, ministre – le mandat de négociation soit rendu public, devait, après sa mise en application provisoire en 2017, être ratifié par les Parlements nationaux.

que vous aviez peur de perdre le vote, comme aujourd’hui. Voilà la réalité ! Monsieur le ministre, n’ayez pas peur. Le débat argumenté et le vote sont la base de la démocratie.

qui instaure une concurrence déloyale pour nos agriculteurs, car les clauses miroirs, malgré vos mensonges, ne figurent pas dans les 2 344 pages du traité et ne sont aujourd’hui qu’un mirage. C’est un traité qui met en place les tribunaux arbitraux privés, juridictions supranationales devant lesquelles les multinationales pourront faire condamner les États si elles considèrent que les lois ont un impact négatif sur leurs investissements.

ci n’aura été possible que parce que nous avons proposé l’examen de ce texte et que, malgré les multiples pressions pour nous faire reculer, voire échouer, nous avons repris la main collectivement sur l’exécutif, qui voulait, jusqu’il y a encore quelques jours, retirer le texte de l’ordre du jour. et Écologiste – Kanaky, qui n’a que deux niches par an, a fait le choix d’inscrire à l’ordre du jour un texte avec lequel il est en désaccord, prenant le risque prenant le risque – je le redis – que le vote final soit contraire à notre position, à nos combats et à notre vision de la mondialisation. Nous l’avons fait, car nos institutions comptent deux chambres, dont le Sénat, et parce qu’il est temps que le processus démocratique soit enfin respecté et complet. Et nous l’avons fait, car il est temps que ces traités de libre échange qui ne sont débattus qu’à huis

Il se murmure déjà, dans les couloirs feutrés des ministères, que vous envisagez de ne pas transmettre le texte à l’Assemblée nationale pour éviter un nouveau débat. Est ce vrai ? Ce n’est j’espère que, ensemble, quel que soit notre vote, nous refuserons ce nouveau déni démocratique. J’ose même parler de « coup de force » ! Monsieur le ministre, vous devez vous engager, dès maintenant, avant le vote,…

s’il avait lieu, s’apparenterait à un nouveau 4 février 2008, jour où le Congrès a ratifié le traité de Lisbonne, contrevenant ainsi au vote populaire de 2005, défavorable au traité constitutionnel. Monsieur le ministre, j’ai une dernière chose

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, enfin ! Enfin, nous allons pouvoir nous prononcer

économique, depuis 2017, les exportations françaises vers le Canada ont augmenté de 33 %, mais les importations ont augmenté de 35 %, pour un effet neutre,

Alors que l’Europe travaille à la diversification de ses sources d’approvisionnement, les industries canadiennes de l’aluminium, du fer, du nickel et du cuivre profitent de la suppression des barrières tarifaires. Il est indéniable que cela permet à l’Union européenne de moins dépendre des marchés russe et chinois. Parlons maintenant de ce qui fâche. Les concessions de la Commission européenne sont en complète contradiction avec le Pacte vert. Ainsi, le Ceta s’accommode de ce qui constitue plusieurs sujets de préoccupation majeurs pour notre agriculture les protéines animales transformées, non autorisées en Europe, les farines animales, non autorisées en Europe, ou encore les 41 substances actives phytosanitaires, non autorisées en Europe.

l’interdiction de l’importation d’animaux nourris aux antibiotiques simulateurs de croissance, il faut se contenter, pour toute garantie, d’une attestation sur l’honneur du vétérinaire, sans contrôle lié. alors que nous traversons une crise agricole sans précédent et que les clauses miroirs ont été l’une des revendications des filières, notamment celle de la viande, comment pouvez vous assumer de telles importations quand tout le monde sait que les contrôles sont impossibles

Comme notre collègue Annick Girardin l’a souligné lors de la séance de questions au Gouvernement du 6 mars dernier, l’article 1.3 du Ceta reconnaît explicitement la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental du Canada, tels qu’ils sont définis dans le droit interne canadien. aucune disposition équivalente n’existe concernant la ZEE et le plateau continental des États membres de l’Union européenne, l’absence de toute réserve ou de déclaration interprétative risquerait, à l’évidence, de constituer un abandon de prétention française légitime dans la zone,

savez bien que, dans un contexte exacerbé de mal être des agriculteurs et de forte pression sociétale, ce texte ne fera pas l’unanimité. Il faut avoir le courage de déplaire à certains pour répondre à des enjeux plus élevés, qu’ils soient économiques, environnementaux ou de santé publique. Le vigneron que je suis, et dont la filière est bénéficiaire, ne peut accepter qu’un accord génère des gagnants et des perdants. Pour notre souveraineté alimentaire, toutes les filières de notre agriculture doivent être solidaires.

députés ont été houleuses. L’accord était alors encore récent, et nous n’avions pas assez de recul sur l’application provisoire de ses dispositions commerciales, en vigueur depuis septembre 2017. Aujourd’hui, nous disposons d’un premier bilan concret de ces dispositions, sur six ans. N’en déplaise à ses détracteurs, ce bilan est positif pour l’Union européenne et la France, comme l’a rappelé M. le ministre. Le Ceta permet à l’Union européenne de tirer un avantage substantiel de ses relations commerciales avec le Canada. En 2018, l’Union bénéficiait déjà d’un excédent cumulé sur l’exportation de ses biens et de ses services vers le Canada de l’ordre de 19 milliards d’euros. La fluidité et l’équilibre de ces échanges sont dus à l’abaissement et à la suppression de 98 % des barrières tarifaires entre l’Union européenne et le Canada. Cette réduction massive des droits de douane favorise l’accès des produits français sur le marché canadien, tout en renforçant leur compétitivité. C’est un réel avantage pour les produits français, dont la population canadienne raffole. À titre d’exemple, la filière viticole, fleuron du patrimoine français, a bénéficié d’une suppression des droits de douane sur les produits qu’elle exporte vers le Canada, sachant que ce pays est notre huitième client mondial pour l’importation de nos vins et le septième pour l’importation de nos spiritueux. Autre exemple qui illustre la réussite du Ceta pour notre économie nationale, l’export des fromages a augmenté de 60 % entre 2016 et 2022. L’excédent commercial des produits laitiers a progressé de 23 millions d’euros entre 2017 et 2023. La conclusion que nous pouvons tirer de ces chiffres est aussi simple que positive : le Ceta offre, depuis 2017, une multitude d’avantages commerciaux tant pour l’Union européenne que pour la France. Les exportations françaises vers le Canada ont progressé de 1 milliard d’euros entre 2017 et 2023, ce qui représente une hausse de 33 %. Nos exportations de services ont, quant à elles, augmenté de 71 % entre 2017 et 2022. Je veux, par ailleurs, insister sur le fait que le Ceta n’est pas un accord de libre échange traditionnel : c’est un accord dit « de nouvelle génération », qui permet aux entreprises françaises de participer de manière accrue au marché public canadien. Il contribue également à l’augmentation des investissements bilatéraux. Il favorise la coopération entre l’Union européenne et le Canada en matière de normes et de régulations. C’est, en somme, un accord essentiel pour la bonne santé économique et commerciale de ses parties prenantes. Malgré cela, certains représentants des filières agricoles et agroalimentaires sont inquiets des conséquences du Ceta. Ces inquiétudes sont partagées par une majorité d’entre vous,

Le Ceta s’est révélé être largement favorable à nos agriculteurs. L’excédent des filières agricoles et agroalimentaires a été multiplié par trois depuis 2017.

de nos débats, on entendait dire que le marché français allait être envahi de bœuf canadien. Pour l’année 2023, la quantité de viande bovine importée sur notre sol depuis le Canada correspond à 0,0034 % de la consommation française. Ce chiffre est très faible, car nous n’importons que des produits satisfaisant à nos exigences sanitaires. Nous écartons ainsi toute importation de viandes traitées aux hormones de croissance, interdites dans l’Union européenne. Si les produits que nous importons ne sont pas conformes aux mêmes normes que celles que respectent nos agriculteurs, nos éleveurs et nos producteurs, ils n’entrent pas sur notre territoire. Je tiens aussi à répondre à celles et ceux qui s’inquiètent des potentielles conséquences négatives du Ceta sur l’environnement. En 2022, l’Union européenne a adopté une nouvelle approche favorisant l’intégration de la durabilité dans les accords commerciaux européens. Elle vise notamment à élever l’accord de Paris au rang d’élément essentiel des futurs accords de commerce de l’Union européenne, au même titre que le respect

En novembre dernier, les deux parties prenantes ont créé l’Alliance verte, pour intensifier la coopération sur des sujets tels que le climat, l’énergie et l’océan. d’avancer dans la bonne direction, d’autant que nous sommes entourés de pays et de personnalités climatosceptiques qui voudraient revenir sur l’accord de Paris de 2015. En outre, quinze des trente matières premières critiques essentielles à notre transition écologique se trouvent au Canada, premier producteur de potasse et deuxième producteur d’uranium au monde. Grâce au partenariat que nous avons signé avec le Canada en septembre 2023,

Nous examinons aujourd’hui le présent projet de loi dans un contexte parlementaire un peu spécial, après plusieurs semaines de crise agricole. Durant cette période, partout en Europe, les agriculteurs ont exprimé deux principales revendications pouvoir vivre dignement de leur métier, de leur travail, d’une part, et ne plus subir une concurrence déloyale des produits exportés à bas coût grâce aux traités de libre échange, d’autre part. L’accord économique et commercial entre l’Union européenne et le Canada a directement trait à ces deux sujets.

décide de recourir aux quotas négociés dans le cadre du Ceta. C’est pour ces filières que la question de la concurrence déloyale se pose au premier chef. Pour nos agriculteurs et pour notre sécurité alimentaire, nous ne pouvons pas accepter du bœuf nourri à la farine d’origine animale et élevé aux hormones de croissance. Nous ne pouvons pas tolérer

Derrière ces mesures de protection des agriculteurs et des consommateurs, c’est la question du modèle agricole que nous voulons pour l’Europe qui se pose. Malheureusement, depuis l’entrée en vigueur provisoire du Ceta, le Canada a cherché à plusieurs reprises à affaiblir la législation européenne en matière agricole, que ce soit en contestant l’interdiction de certains produits phytosanitaires ou en cherchant à obtenir des dérogations pour l’exportation de viande bovine. Ce lobbying, rendu possible par les forums réglementaires prévus par l’accord, n’est pas acceptable et n’est pas à la hauteur des ambitions environnementales et climatiques que nous devons défendre. Il est également important de rappeler que le Ceta a déstabilisé la filière laitière canadienne, dont l’organisation reposait encore sur des quotas afin d’assurer une juste rémunération des agriculteurs. Les effets de cet accord sont donc dommageables pour les paysans des deux côtés de l’océan Atlantique. Plus largement, ce traité de libre échange a surtout permis une augmentation des échanges de produits fortement carbonés, ce qui est bien sûr intolérable pour un accord dit de « nouvelle génération

partagent une histoire, une culture et une langue commune. C’est en raison de cette amitié, loin des caricatures, que nous ne pouvons pas tout accepter,

halte aux caricatures, place à la cohérence ! Mes chers collègues, la vérité se situe entre les deux : je crois qu’un équilibre peut et doit être trouvé, car il ne s’agit pas ici de remettre en cause le libre échange. Le président de notre groupe, Bruno Retailleau, l’a rappelé : nous croyons en la liberté et dans le commerce comme potentielles sources de prospérité des peuples.

Il est incohérent d’imposer des normes de plus en plus contraignantes à nos producteurs, en les exposant toujours plus à des concurrents qui ne respectent pas les mêmes règles que les nôtres. Comment pourrions nous continuer à prétendre que nous défendons l’environnement, que nous voulons une production raisonnée, plus respectueuse des équilibres écologiques si, après avoir rendu la vie impossible aux paysans

avec lequel nous partageons une histoire, des intérêts convergents et, surtout, des perspectives d’avenir. Eh oui ! Depuis sept ans, nous constatons que les filières fromages, vins et spiritueux, ou encore

aux producteurs européens pour préserver la santé de nos ressortissants. Le Canada – et c’est son droit – utilise quarante molécules de pesticides interdits dans l’Union européenne. Il cherche avec insistance à utiliser de l’acide peracétique – interdit en France – pour décontaminer les carcasses

le droit des gouvernements à réguler dans l’intérêt général et à protéger la santé publique et l’environnement. L’avenir du projet européen et du libre commerce passe par des traités équilibrés, respectueux des normes et des priorités européennes. Monsieur le ministre, la politique commerciale européenne ne doit plus se résumer à traiter telle ou telle filière comme une monnaie d’échange, au mépris des règles que l’Europe impose sur son propre marché intérieur. Plus encore, l’Union européenne doit rester souveraine et décider des règles qu’elle applique sur son territoire, sans être empêchée par des accords ou menacée par des multinationales. Au sein de l’Union Centriste, chacun votera selon ses convictions, mais nous souhaitons tous développer un partenariat commercial juste et équilibré avec ce pays frère qu’est le Canada. Il suffit

vigueur de cet accord, en septembre 2017, a entraîné la levée immédiate de près de 98 % des barrières tarifaires pesant sur les échanges entre l’Union européenne et le Canada. Le secteur agricole a donc connu une libéralisation des échanges, marquée par la disparition programmée de près de 94 % des droits de douane. Les produits agricoles et ceux qui sont issus de l’industrie agroalimentaire sont en effet au cœur des échanges entre l’Union européenne et le Canada. Le Ceta s’est révélé être bénéfique pour quelques produits agricoles français qui ont largement pénétré le marché canadien.

Sénatrice de la Manche, je me dois de rappeler ici que le lait est le premier secteur de l’économie agricole normande, avec près de 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le produit laitier spécifique à la Normandie est bien sûr le camembert. La région fabrique 83 % des camemberts français, et nos laiteries produisent près de 43 % des fromages frais français. La filière laitière est aussi le premier pourvoyeur d’emplois du secteur agroalimentaire.

recensées. Malgré ces arguments, une large majorité des acteurs du monde agricole s’oppose à la ratification de ce traité, car elle estime que certaines filières ne bénéficient pas des garanties nécessaires. En effet, les différences de conditions d’élevage entre nos deux pays et la faiblesse des contrôles sanitaires qui devraient être effectués par chaque État membre peuvent favoriser l’importation de viande bovine élevée aux antibiotiques et aux accélérateurs de croissance. Cela reviendrait à proposer aux consommateurs français et européens des produits bien en deçà de nos standards, à bas coût, qui mettraient en péril la filière bovine française.

En effet, le Canada est un partenaire incontournable pour l’économie européenne : il fournit quinze des trente métaux et minéraux considérés comme critiques, tels que l’aluminium, le nickel, le cuivre, le plomb et le zinc.

l’accord commercial avec le Canada représente donc une occasion de développer les échanges commerciaux avec un État dont les standards sociaux et environnementaux sont proches de ceux de la France.

Oui, nous sommes pour le libre échange avec nos amis canadiens, mais cela suppose, comme l’a dit notre collègue Valérie Boyer, des échanges libres et équilibrés. C’est pourquoi il est nécessaire de supprimer l’article 1 de ce projet de loi.

Ces deux articles – ces deux accords – sont parfois présentés comme les versants économique et politique d’un même rapprochement entre l’Union européenne et le Canada. Or il s’agit bien de deux accords distincts. Ainsi, si dix parlements nationaux n’ont pas ratifié le Ceta, seuls trois États, dont la France, n’ont pas approuvé l’accord de partenariat stratégique, ce qui est bien la preuve que les deux sont dissociables. C’est aussi la aussi la preuve que l’article 1 relatif au Ceta et l’article 2 relatif à l’accord de partenariat stratégique peuvent faire l’objet de votes opposés. J’ajoute, car cette question a été posée en commission, que la mise en place d’un mécanisme juridictionnel destiné au règlement des différends entre investisseurs

Mes chers collègues, si certains d’entre nous sont en désaccord avec le contenu du Ceta, en raison notamment des risques qu’il fait peser sur le monde agricole, il me semble que nous ne pouvons qu’être favorables à un resserrement des liens politiques avec le Canada,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de nous prononcer sur cet article, il est important de rappeler

mais ce traité, amorcé sous la présidence de Nicolas Sarkozy, voulu par la présidence de François Hollande, entré en vigueur en 2017, suscite aujourd’hui beaucoup de crispations, notamment au sein de plusieurs filières agricoles, et de l’incompréhension chez certains d’entre nous. En effet, en sept ans,

Monsieur le ministre, comme vous, nous pensons que notre politique commerciale doit contribuer à accroître la résilience de l’Union européenne dans les domaines climatique et sanitaire, qu’il faut renforcer la cohérence entre notre stratégie commerciale et notre engagement en faveur du développement durable et du climat. C’est pourquoi nous sommes opposés à la ratification de cet accord, qui est en contradiction avec les objectifs que vous avez évoqués à plusieurs reprises depuis 2020. À l’heure où la biodiversité s’effondre, où le climat se dérègle, où les températures augmentent, mettant en difficulté notre agriculture, comment croire que la multiplication des échanges puisse être une solution viable ? Comment croire que l’augmentation des importations de pétrole de schiste ou de ses produits dérivés puisse être une bonne nouvelle pour l’environnement ? Pourquoi minimiser les menaces pesant sur la filière bovine française et la mise en concurrence des éleveurs qui ne sont pas soumis aux mêmes normes ? Malgré vos discours, monsieur le ministre, la réalité est têtue. Les normes qui s’appliquent à l’Union européenne ne sont pas respectées par nos partenaires canadiens

ces raisons, nous sommes contre cet accord et demandons la suppression de l’article 1. La